Nous reprenons la discussion de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice et de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice. Dans la suite de la discussion générale commune, la parole est à M. Yves Détraigne.

La justice va mal. Ses délais ne cessent de s'allonger. En dix ans, ils sont passés de sept mois et demi à près d'un an pour les tribunaux de grande instance. Dans le même temps, le stock d'affaires en attente d'être jugées a augmenté de plus de 25 % pour les juridictions civiles.

le constat sévère que nous avons collectivement dressé lors des travaux de la mission d'information sur le redressement de la justice. Le constat est sévère, mais, pis encore, il n'est pas une surprise, en tout cas pas pour ceux qui, comme moi, s'intéressent depuis des années aux moyens dont dispose la justice. Depuis des années, en effet, dans le cadre de l'examen des crédits de la mission « Justice », j'alerte la Haute Assemblée et les gouvernements successifs sur l'état de nos tribunaux, sur l'impossibilité pour certaines juridictions de régler les frais de justice avant même que la moitié de l'année soit écoulée, sur les vacances de postes, etc. Nous ne pouvons plus attendre. C'est pour cela que je salue l'inscription à notre ordre du jour de ces deux textes. Je salue également l'important travail réalisé dans le cadre de la mission d'information et sur les deux propositions de loi par les corapporteurs, Jacques Bigot et François-Noël Buffet. Ils ont su préserver l'esprit général de la mission d'information tout en apportant certaines modifications afin de

pour une fois, elle ne dissocie pas les aspects budgétaires du fond de la réforme. Les deux textes apportent des évolutions importantes, aussi bien en matière d'organisation judiciaire que sur le statut et l'organisation de la magistrature. Dans les deux cas, les évolutions proposées sont financées. Ils ne font pas l'impasse sur ce qu'on pourrait appeler les serpents de mer qui hantent la place Vendôme. Je pense, par exemple, à l'aide juridictionnelle et à son financement. Nous vous proposons de rétablir la contribution pour l'aide juridique supprimée par la loi de finances pour 2014. Cette contribution apporte une réponse simple et efficace au besoin de financement de l'aide juridictionnelle, pour un coût modique pour le justiciable. Même si cette mesure ne résoudra pas à elle seule les questions posées par l'aide juridictionnelle, elle devrait néanmoins générer plus de 50 millions d'euros chaque année. Autre sujet très sensible : l'organisation judiciaire. Chacun se souvient des débats enflammés suscités par la réforme Dati en 2007-2008. Aujourd'hui, la commission des lois opte pour la création d'un tribunal départemental unique de première instance, regroupant le tribunal de grande instance et les tribunaux d'instance de son ressort.

Pour autant, plusieurs de nos collègues ont émis en commission un certain nombre de craintes. C'est pourquoi Sophie Joissains a souhaité que cette innovation soit d'abord expérimentée dans quelques départements pendant trois ans, avant d'être généralisée à l'ensemble du territoire. Elle proposera un amendement en ce sens. Concernant la magistrature, de nombreuses évolutions ont eu lieu récemment avec la loi organique du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats Ce texte a notamment permis d'ouvrir davantage le recrutement et diversifier le corps de la magistrature ; c'est une avancée. Pour autant, il restait encore de nombreuses pistes d'évolutions à explorer, notamment en matière de gestion des ressources humaines. Une question importante est celle des postes offerts à la sortie de l'École nationale de la magistrature. Comme le mettait déjà en évidence en 1994 Jean-Jacques Hyest, à l'époque député chargé par le Premier ministre d'établir un rapport sur la formation professionnelle des magistrats et des avocats, « un magistrat sortant de l'ENM va immédiatement, dans la majorité des cas, assumer les responsabilités de juge d'instruction, de juge des enfants, de juge d'application des peines ... il continuera d'exercer des fonctions de même type avec des responsabilités quasiment identiques ». Depuis lors, cette situation, en dépit de critiques récurrentes, n'a guère évolué. Il apparaît contre-productif de confier à des débutants des postes peu attractifs en raison d'un contexte difficile- nature, localisation du poste ou autre motif -et susceptible d'engendrer à terme un certain découragement. Cela alimente le phénomène, relevé par la mission d'information, de turn-over important sur certains postes, où les magistrats, à peine arrivés, demandent leur mutation. Au contraire, il faudrait nommer les jeunes magistrats à des postes adaptés à leurs capacités. Aujourd'hui, ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Les pistes de réflexion sur ce sujet sont nombreuses. On peut se rappeler de ce que préconisait notre regretté collègue Pierre Fauchon dans un rapport datant de 2006 qui prévoyait l'instauration d'une période de probation d'au moins deux ans au sortir de l'ENM, le magistrat débutant étant alors dénommé « magistrat référendaire Sans aller jusque-là, je me félicite du maintien dans le texte des dispositions prévues aux articles 4 et 7. Elles créeront de nouvelles possibilités de collaboration entre magistrats du siège pour le traitement des décisions complexes. Elles permettront notamment au magistrat chargé d'une affaire de bénéficier d'un renfort précieux pour préparer sa décision et au jeune magistrat de perfectionner sa formation. Plus fondamentalement, il me semble que le critère déterminant pour l'affectation de magistrats sortis d'école devrait être l'affectation dans des formations systématiquement collégiales, à l'exclusion de toute affectation sur un poste à juge unique, s'il s'agit de fonctions spécialisées comme juge d'instruction ou juges des enfants. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, madame la garde des sceaux, le groupe Union Centriste partage les objectifs de ces deux textes d'initiative parlementaire Il n'est plus temps de commander de nouveaux rapports d'information- j'ai participé à cela - : il faut agir ! J'espère, madame la garde des sceaux, que le Gouvernement entendra la voix constructive du Sénat, dans l'intérêt des acteurs du monde judiciaire, mais aussi et surtout dans l'intérêt de nos concitoyens.

Cette situation résulte de divers facteurs : accroissement du recours à la justice par nos concitoyens, réformes pénales successives n'ayant pas permis de désengorger des prisons surpeuplées, insuffisance des moyens affectés à la justice. Dans ce contexte, en tant que rapporteur spécial des crédits de la mission « Justice », je souscris bien sûr à l'idée que le ministère de la justice doit être considéré comme prioritaire et, à ce titre, voir son budget augmenter quand des économies sont demandées à d'autres. Pour aller plus loin, la commission des lois propose notamment une trajectoire pluriannuelle d'augmentation des crédits et des emplois de la mission « Justice » sur cinq ans. Une telle programmation est attendue par le monde judiciaire : source de prévisibilité, elle serait le gage d'une meilleure gestion,

En effet, des réformes sont attendues en matière d'organisation, mais aussi de procédures, de délais de jugement, de dématérialisation et d'informatisation, d'accessibilité de la justice. Évaluer l'efficacité des dispositifs et des réformes : c'est sous cette condition qu'une augmentation des moyens est envisageable. Si le budget du ministère de la justice s'inscrit, ces dernières années, dans une phase de rattrapage, il convient de préparer une seconde phase, susceptible de permettre la réalisation d'économies. Je pense en outre que l'existence d'un budget pluriannuel de la justice constitue sans nul doute un outil au service du ministre de la justice, notamment lors des arbitrages budgétaires. Toutefois, je souhaiterais formuler deux remarques sur la trajectoire des crédits proposée à l'article 2 de la proposition de loi. Il est préférable de prévoir les moyens supplémentaires pour une politique publique prioritaire en examinant, dans le même temps, les modalités de leur financement et le cadre global dans lequel ils s'inscrivent ; je pense en particulier à nos engagements européens. Ce sera l'objet du débat que nous aurons dès la semaine prochaine sur le projet de loi de programmation des finances publiques. Les trajectoires proposées pour le budget de la justice par le Gouvernement et la proposition de loi ne sont pas identiques. L'article 2 de la proposition de loi prévoit, pour la période entre 2018 et 2022, une augmentation plus de 25 % des crédits de la mission. L'horizon du Gouvernement s'arrête à 2020. Le projet de loi de finances pour 2018 attribue 6 millions d'euros de plus à la mission « Justice » que la proposition de loi. Entre 2018 et 2020, le projet du Gouvernement accroît les moyens de la justice de 9,6 %, contre 7,9 % dans la proposition de loi. Par ailleurs, contrairement à la méthodologie des lois de programmation des finances publiques, la trajectoire de la commission des lois intègre l'évolution de l'inflation et de la contribution au compte d'affectation spéciale « Pensions ». La dynamique propre de ces variables pourrait absorber une partie de l'effort en faveur des moyens de la justice.

lois ! Je terminerai par quelques remarques concernant l'article 1 de la proposition de loi organique, qui vise à exonérer de gels et d'annulations les crédits des juridictions judiciaires et du Conseil supérieur de la magistrature. Le caractère constitutionnel d'une telle disposition n'est pas certain, comme le soulignent justement les rapporteurs : la régulation budgétaire appartient d'abord au Gouvernement, même si le Parlement peut l'encadrer. Il le fait d'ailleurs dans les lois de programmation des finances publiques. Surtout, les annulations comme les mises en réserve permettent de piloter les dépenses pour tenir compte des évolutions de la conjoncture et des urgences auxquelles il faut faire face en cours d'année, tout en évitant de dégrader le déficit de l'État.

: j'imagine déjà les demandes de même nature qui ne manqueraient pas d'émaner d'autres secteurs de l'action publique ! C'est pourquoi je ne voterai pas l'article 1 de la proposition de loi organique. Sous ces réserves, qui portent

titre, le mot d'ordre qui a guidé la rédaction de ce rapport d'information et des propositions de loi qui en résultent. Nous les examinons ce soir avec beaucoup de volonté,

Le groupe socialiste et républicain accueille favorablement, en effet, les propositions de loi tant elles s'inscrivent dans la continuité et prolongent l'action du dernier quinquennat pour améliorer le fonctionnement de la justice, à partir d'un constat sans concession que nous pourrions résumer ainsi : nous n'avons pas été collectivement à la hauteur des enjeux rencontrés par la justice de notre pays. Plusieurs questions sont posées par ces textes comment fait-on pour donner envie aux jeunes magistrats de rester en poste dans des juridictions difficiles ? Comment assurer l'effectivité de l'exécution des peines ? Comment faire en sorte que les moyens de la justice soient en corrélation avec la mission de service public dont elle

constructives. Malgré une augmentation régulière du budget de la justice, ce dernier, cela a été dit à de nombreuses reprises, demeure insuffisant. Il faut continuer et amplifier la dynamique vertueuse enclenchée, notamment sous le précédent quinquennat, qui a permis de nombreuses avancées : l'augmentation de près de 15 % du budget en cinq ans ; la création de 6 000 postes dans la justice, dont 1 714 dans les services judiciaires

seul critère qui nous permettra de mettre en cohérence l'ambition partagée par les membres de cette assemblée avec des réalisations concrètes. Sur ce point,

Ce combat, c'est aussi un combat pour avoir les moyens de mettre en oeuvre les sanctions, pour que la peine soit efficace. Il faut cesser d'avoir des peines d'emprisonnement prononcées qui ne sont pas exécutées. Les Français ne le comprennent pas et y voient un signe de faiblesse de notre République. Il faut aussi un système pénitentiaire qui prévienne la récidive, l'augmentation de ses capacités. Ces cinq dernières années, 8 000 nouvelles places de prison ont été créées afin de lutter contre la surpopulation carcérale et tendre vers l'encellulement individuel. Ces textes continuent le travail mené, et nous les approuvons. Un dispositif comme celui de la contrainte pénale, par exemple, pourrait bénéficier d'une meilleure mise en oeuvre avec l'augmentation souhaitée des moyens de la justice. Je sais que la majorité au Sénat l'a remise en cause dans une précédente proposition de loi. En cohérence avec les ambitions affichées ici, je suis convaincu que cette mesure continuera à participer à une justice plus efficace. ! Cela Cela serait logique, car la proposition de loi ordinaire, comme la loi du 1 août 2014, affirme notre volonté de renforcer l'individualisation de la réponse pénale, qui permet d'apporter une réponse à l'acte posé en adéquation avec sa gravité et avec le profil de l'intéressé. Cette loi,

une lutte sans merci face à la récidive, principale source de mécontentement de nos concitoyens. Ces textes respectent aussi l'esprit de la loi de modernisation de la justice du XXI siècle, avec, par exemple, la modernisation du service public de la justice, par l'innovation et la maîtrise de la révolution numérique, ou encore l'amélioration de l'organisation de la justice à proprement parler. La proposition de loi reprend ainsi un point très intéressant du rapport de la mission d'information : la création d'un tribunal départemental de première instance, venant remplacer les tribunaux d'instance et les tribunaux de grande instance sans remettre en cause la carte judiciaire. Comme la loi de modernisation de la justice du XXIsiècle, elle s'inscrit dans la perspective de décharger le juge de certaines tâches, en renforçant notamment le poids des conciliateurs de justice et en lui permettant de se reposer davantage sur des juristes assistants. La proposition de loi organique, qui vise à stabiliser la nomination des magistrats, va également dans le bon sens. Une trop grande mobilité des magistrats peut être préjudiciable à certaines juridictions. Qu'ils restent au moins trois ans dans leur affectation, quatre dans le cas des fonctions spécialisées, et qu'une certaine souplesse soit laissée au Conseil supérieur de la magistrature participe à la bonne organisation de la justice. de la justice. Certes, tous les chantiers de la justice ne sont pas résolus ici, et c'est bien normal. Je pense notamment à la réforme du statut du parquet. On ne peut que regretter que les conditions n'aient pas été réunies précédemment pour la mener à son terme. Je profite donc de votre présence, madame la garde des sceaux, pour passer le message et espérer que nous avancerons sur ce sujet. Par ailleurs, je suis heureux que l'examen de ces textes par la chambre haute se télescope, si je puis dire, avec les annonces que vous avez faites lors du conseil des ministres du 4 octobre dernier et que vous avez rappelées devant notre assemblée. Ainsi, vous allez lancer cinq grands chantiers qui visent à transformer en profondeur deux aspects majeurs de la question qui nous occupe : l'amélioration du fonctionnement quotidien de la justice et l'efficacité des peines. Si je ne peux que m'en féliciter, tant ces annonces font écho au travail que nous réalisons aujourd'hui, j'exprime pourtant un regret. Pourquoi donc se cantonner aux annonces quand l'urgence est manifeste ? Le diagnostic est connu de tous. Le temps de la poursuite de l'action est venu ; c'est un besoin impérieux. Aussi j'espère que la discussion que nous allons avoir aujourd'hui sera féconde et, pourquoi pas, garde des sceaux, aider ces textes à prospérer dans la suite de la navette parlementaire ... Vous me répondrez probablement, vous l'avez d'ailleurs déjà presque fait, que ces sujets méritent une importante concertation et que vous nous proposerez bientôt un projet de loi, ce à quoi je me permettrai d'opposer l'urgence évoquée précédemment. Vous avez annoncé un « véritable plan d'action », qui « doit être élaboré dans des délais rapprochés pour que les réformes nécessaires puissent intervenir rapidement ». Nous vous offrons ici un support qui permettrait de raccourcir ces délais. C'est pourquoi, madame la garde des sceaux, j'invoque la nécessité d'aller dès à présent encore plus loin, plus vite, plus fort. Vous le voyez, je le répète, le groupe socialiste et républicain porte un regard bienveillant sur les présentes propositions de loi. Des améliorations ont été apportées en commission ; je pense notamment à la suppression de la condamnation à une amende civile de 10 000 euros en cas d'appel ou de pourvoi jugé dilatoire ou abusif en matière pénale. C'était un obstacle à l'accès à la justice et une atteinte aux règles du procès équitable. C'est une bonne chose que la commission et ses rapporteurs, que je salue, aient accepté à deux reprises de prendre en considération la proposition du groupe socialiste et républicain. Je remercie Je remercie également la commission d'avoir, grâce à un débat lancé par le dépôt d'un amendement que j'ai défendu au nom du groupe socialiste et républicain, acté la mise en place d'un groupe de travail sur la présomption irréfragable de non-consentement des mineurs à un acte de pénétration sexuelle. Je me permets cette digression, car, si le lien avec le texte est certes ténu, cette question relève également de l'amélioration de la justice. Nous comblerions ici un vide juridique qu'une actualité judiciaire douloureuse nous a rappelé il y a quelque temps. Malgré ces points d'accord, nous avons plusieurs points de divergence avec la proposition de loi ordinaire. La réinstauration d'une contribution à l'aide juridictionnelle et l'inscription dans la loi du principe d'une consultation juridique préalable à la demande d'aide juridictionnelle afin de vérifier que l'action envisagée ne paraît pas manifestement irrecevable

Par ailleurs, baisser les seuils d'aménagement de peine ou étendre le suivi socio-judiciaire ne nous semble pas cohérent avec la volonté de rendre les peines plus efficaces et donc avec l'esprit du texte. Je développerai ces points plus longuement lors de l'examen des amendements,

un amendement sur ce sujet. Pour conclure, je suis heureux que nous oeuvrions ensemble pour surmonter les obstacles importants qui s'offrent à nous et que nous fassions preuve d'intelligence collective pour conforter la confiance des Français en leur justice. Nous ne pourrons pas être d'accord sur tout, c'est l'essence même de la démocratie, mais il convient de nous rassembler pour avancer sur les sujets qui sont la clé de voûte de la République. J'en appelle donc encore une fois à vous, madame la garde rejoignez-nous pour qu'ensemble nous accélérions un processus qui sera porteur de progrès supplémentaires pour tous nos concitoyens et donnera l'image d'une République ferme et généreuse.

Ce constat, c'est celui de la dégradation constante de la justice, du besoin de réformes structurelles profondes, de nature à améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'institution judiciaire, indépendamment ou, en tout cas, en complément d'un redressement significatif et durable de ses moyens. Dans ce domaine de votre ministère, comme dans d'autres, il y a sans doute une méprise ou tout au moins une insuffisance qui demeure et qui consiste à considérer les enjeux d'un bon

: la maîtrise des délais. Question essentielle en effet pour une bonne justice que celle des délais de jugement. De ce point de vue, le renforcement des moyens humains dans les juridictions, par l'augmentation des crédits de 5 % par an, l'amélioration des outils informatiques par la sécurisation juridique de l'des décisions,

mobilité. Troisième objectif : une plus grande proximité de la justice pour le justiciable, tout au moins pour les litiges de la vie courante. Cela passe par une organisation territoriale de proximité, c'est-à-dire un tribunal départemental unique de première instance avec des chambres détachées par la création d'un tribunal des affaires économiques, avec l'extension de la compétence du tribunal de commerce aux agriculteurs, professions libérales et associations un assouplissement de l'organisation prud'homale, avec une composition des sections variable, en fonction du contentieux ; enfin, par la révision du financement structurel de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire le rétablissement du droit de timbre et la consultation obligatoire d'un avocat avant toute demande d'aide.

au XIV siècle d'un bon ou d'un mauvais gouvernement, c'est-à-dire d'une justice qui affirme et garantisse le droit des plus faibles.

vingt-huit articles, la proposition de loi organique en compte quinze. Depuis de nombreuses années, nous assistons à une dégradation constante de la justice, malgré une progression des crédits dans chaque loi de finances. En 2002, les crédits de la mission « Justice » s'élevaient à 4,5 milliards d'euros ; en 2017, ils atteignent 8,5 milliards

On notera quatre priorités. La première est la maîtrise des délais grâce à un renforcement des moyens humains, tout en incitant à la conciliation. deuxième est l'amélioration de la qualité des décisions, notamment, comme cela a été rappelé par plusieurs de nos collègues, en remédiant au problème de la mobilité des magistrats. troisième est le renforcement de la proximité de la justice pour le justiciable. Il est en effet indispensable de disposer d'une organisation territoriale de proximité : tribunal départemental unique, mise en place d'un tribunal des affaires économiques, extension de la compétence du tribunal de commerce aux agriculteurs, professions libérales et associations. Cette ouverture aux acteurs économiques est tout à fait fondamentale. La quatrième priorité concerne l'amélioration de l'effectivité afin de réduire le risque de récidive. Il en résulte une augmentation des capacités pénitentiaires parallèlement à un renforcement des moyens humains du personnel qui oeuvre dans les prisons et exerce des métiers particulièrement difficiles. Nous sommes conscients que la tâche est immense. Sur le terrain, dans nos départements respectifs-

que votre première intervention sur l'article 1 soit pour contester l'affirmation en vertu de laquelle il ne faudrait pas qu'il y ait des gels de crédits en cours d'année.

ne signifie pas que le Gouvernement n'est pas décidé à se battre pour que les crédits du budget de la justice soient en augmentation.

de l'augmentation du budget ni même sur la nécessité, que nous partageons avec la commission et vous-même, d'avoir des crédits en augmentation pour les services judiciaires. Je veux simplement dire que je m'interroge sur la constitutionnalité d'une disposition qui prévoit de restreindre la compétence et les prérogatives du Gouvernement en matière d'exécution budgétaire.

Madame la garde des sceaux, je ne veux pas prolonger excessivement cet échange : nous avons bien compris que le Gouvernement ne souhaitait pas que soit

: La parole est à Mme Josiane Costes. Cet amendement de suppression vise à marquer notre désaccord sur la répartition des crédits proposée. Il s'agit non pas de mettre en cause la sincérité de la programmation, mais plutôt de souligner la différence de nos approches respectives concernant le redressement de la justice. Nous aurions souhaité que l'effort en direction de l'autorité judiciaire soit plus important. Une fois encore, le programme « Administration pénitentiaire » absorbe une grande partie des crédits. En effet, sur un total de 2,17 milliards de progression de l'ensemble de la mission « Justice 1,59 milliard est fléché vers l'administration pénitentiaire, soit trois fois plus que pour le programme « Justice judiciaire ». La surpopulation carcérale et le délabrement de nos prisons sont indéniables. La situation des prisons françaises a d'ailleurs donné lieu à de nombreuses condamnations de l'État devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais la France a également déjà été condamnée pour ses procédures judiciaires trop lentes. Les deux situations sont donc prioritaires. Comme nous l'évoquions précédemment, il nous paraît donc illusoire de vouloir résoudre ces deux problèmes avec le même outil budgétaire, en maintenant une justice de qualité et accessible. Cela nous conduit toujours à arbitrer entre l'un et l'autre : la programmation proposée n'en est qu'une énième démonstration.

Il faut une loi de programmation pour la justice, mais je m'étonne que vous préemptiez ce que décideront celles et ceux qui vous succéderont.

Les rapports de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice permettent de mettre en lumière la sous-dotation structurelle de nos juridictions en effectifs, par comparaison avec les effectifs recensés chez nos voisins européens. En 2014, la France comptait ainsi deux fois moins de juges professionnels que la moyenne européenne, quatre fois moins de procureurs et deux fois moins de non-magistrats. La répartition de l'augmentation des plafonds d'emplois retenue prévoit une hausse d'environ 6 % des effectifs du programme « Justice judiciaire un peu plus de 2 000 personnes, contre une hausse de 21 % pour l'administration pénitentiaire. Cela ne nous semble pas aller dans le sens d'un rattrapage de notre retard au regard de nos voisins européens.

de recrutement consenti en faveur de l'administration pénitentiaire : nous l'avons déjà dit, cela représente 1 500 postes de surveillants en plus. Il s'est également agi d'accompagner l'ouverture de nouveaux établissements pénitentiaires, puisque l'on tient compte de la construction de 15 000 places supplémentaires. Des recrutements significatifs sont également prévus au bénéfice des juridictions. Je voudrais les citer dans le détail : la programmation des emplois vise notamment à combler la vacance de postes de magistrats- 500 postes -et de greffiers- plus de 900 postes sur cinq ans -, mais aussi à prévoir la création de postes de greffiers assistants de magistrats- 100 postes -et de juristes assistants- 300 postes -destinés à renforcer l'équipe du juge, ainsi qu'à accroître les effectifs mis à disposition des chefs de cour et de juridiction, en

L'objectif semble être d'accorder une plus grande place à la conciliation dans l'architecture judiciaire, en permettant au conciliateur de présenter au juge une proposition de règlement du litige et en exploitant si nécessaire la main-d'oeuvre bon marché que constituent les assistants de justice pour s'acquitter de cette fonction. Sur le plan programmatique, cette volonté se traduit donc par le recrutement de 1 200 conciliateurs supplémentaires, en plus des 2 200 existants. Certains se féliciteront du faible coût de la mesure, puisque les conciliateurs sont bénévoles et que les assistants de justice sont rémunérés entre 450 et 500 euros nets mensuels, selon une information publiée sur le site internet du ministère de la justice. Derrière l'économie budgétaire, on peut cependant s'inquiéter du coût caché d'une telle mesure pour le justiciable, pour qui la conciliation pourrait représenter une étape supplémentaire dans un parcours judiciaire déjà long. D'autant que peu d'informations sont disponibles sur l'avenir des conciliations et la satisfaction qu'en tirent les personnes qui y ont recours. À ce propos, la décision des rapporteurs de ne pas conférer à l'accord issu de la conciliation la force exécutoire est une bonne chose. Nous ne sommes pas opposés par principe à la conciliation, bien que ce soit une forme de déjudiciarisation, mais nous souhaiterions disposer de renseignements susceptibles de nous convaincre de son utilité, pour la gestion du flux de contentieux comme pour le justiciable. Tel est l'objet de cet amendement.

des conciliateurs est d'amener les gens à se réconcilier. Ce n'est pas du tout gênant ! Si l'on arrive à décharger les magistrats de ce type de contentieux, ce serait une bonne chose pour la justice. Voilà le motif pour lequel la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

plus considérés, par les nombreuses personnes qu'ils reçoivent chaque semaine dans nos mairies, comme des juges : elles attendent d'eux qu'ils rendent un jugement.

le manque de magistrats. La réalité, mes chers collègues, c'est que la France consacre chaque année 72 euros par habitant à la justice, contre 146 euros en Allemagne et 155 au Royaume-Uni.

des noms des magistrats qui les ont rendus. Le Conseil national des barreaux s'est opposé à l'unanimité à cette anonymisation. De même, le Premier président de la la Cour de cassation et les premiers présidents de cour d'appel se sont prononcés contre cette mesure, qui ferait de la France une exception en Europe, la plaçant aux côtés de la Russie et de la Roumanie en matière de transparence. En outre, la Commission

: La parole est à Mme Josiane Costes. L'objet de cet amendement est de prévoir des obligations légales minimales s'imposant aux sites internet dispensant des informations et des renseignements juridiques, afin qu'elles prennent effet le plus rapidement possible. Il arrive en effet que certains projets de décret se perdent dans la mécanique gouvernementale ... Compte tenu de l'influence de ces informations disponibles en ligne sur les justiciables, apporter cette précision nous semble important. La mobilisation de tous les acteurs du droit est nécessaire pour lutter contre les recours abusifs ou irrecevables et désengorger nos tribunaux. par mes collègues. Quel est l'avis de la commission ?

pouvant découler des dispositions de l'article 7 aux termes desquelles toute personne peut proposer, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne fournissant des prestations d'information juridique ou d'aide à la saisine de juridictions. L'alinéa 3 prévoit que ces sites peuvent proposer des actes d'assistance ou de représentation, à la condition de recourir à un avocat. Nous considérons qu'il sera difficile pour un justiciable de s'assurer qu'un avocat est associé aux actes mentionnés avant de souscrire un contrat un contrat de services, sauf à ce que le nom de l'avocat figure sur le site internet concerné, obligation qui n'est pas prévue par l'article. Ce dispositif est de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des justiciables. En outre, nous estimons que le développement d'une intermédiation de la relation entre justiciable et avocat est de nature à accroître les frais de justice, ce qui ne va pas dans le sens d'une meilleure accessibilité Pour ces raisons, nous souhaitons interdire strictement aux personnes n'exerçant pas la profession d'avocat de proposer des services d'assistance ou de représentation juridique au sens de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971. Quel est l'avis de la commission ?

Il est ainsi prévu d'imposer des règles de déontologie et une obligation d'information du public aux personnes proposant en ligne une assistance juridique ou une aide à la saisine

proposition de loi ne semblent pas avoir d'idée précise des mécanismes qui seraient susceptibles de constituer de véritables garanties en la matière, ce qui nous semble pour le moins inquiétant. ailleurs, comme le souligne le Syndicat de la magistrature, dont nous avons entendu les représentants il y a peu, il semble, monsieur Bas, que vous considériez la résolution de litiges en ligne comme une solution miracle au problème majeur de l'engorgement des juridictions. Nous ne sommes pas contre cette idée ; cela mérite probablement une réflexion approfondie. Toutefois, de notre point de vue, l'objectif doit toujours être de maintenir un accès garanti à tous et gratuit à la justice de notre pays. Or nous parlons ici de services en ligne payants qui créeront, sans nul doute, de nouvelles inégalités entre justiciables. Pour toutes ces raisons, les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste

à encadrer la résolution des litiges en ligne et à instaurer un service public gratuit en ligne d'aide à la résolution amiable des litiges.

Cela illustre la difficulté de nos services à passer des marchés d'équipement informatique et de logiciels à des prix raisonnables. L'alinéa 5 de l'article 8 de la proposition de loi prévoit la création d'un service public gratuit en ligne d'aide à la résolution amiable des conflits. Compte tenu de la forte contrainte budgétaire pesant déjà sur le ministère et de l'obsolescence générale du matériel mis à disposition, cet investissement paraît secondaire. En outre, si l'on considère que le coût de CASSIOPÉE s'élève au total à 142 millions d'euros,

: La parole est à Mme Josiane Costes. Nous avions considéré, dans un premier temps, que l'harmonisation des jurisprudences, la gestion des flux et des stocks de contentieux et l'amélioration de la qualité des décisions relevaient du domaine de la loi. Nos échanges en commission des lois ce matin nous ont convaincus du contraire. Nous retirons donc cet amendement, non sans avoir exprimé l'inquiétude que nous inspirent l'utilisation qui pourrait être faite des données contentieuses mises à disposition du public et le développement possible de ce que l'on appelle la justice prédictive.

près la Cour de cassation donne seulement des avis à la Cour, sans exercer aucune responsabilité en ce qui concerne les décisions juridictionnelles, contrairement à ce que laisse entendre l'exposé des motifs de l'amendement. C'est pourquoi, la mission de tenir les bases de la jurisprudence et de la diffuser incombe au seul service de la documentation, des études et du rapport, dirigé par un président de chambre, composé exclusivement de magistrats du siège et placé sous l'autorité du seul Premier président.

le Premier président et le procureur général veillent à ce que la réutilisation des informations figurant dans les décisions mises à la disposition du public en application de l'article L. 111-13 favorise l'harmonisation des jurisprudences, prévienne le contentieux en matière civile, contribue à améliorer la qualité des décisions de justice et ne porte pas atteinte à la liberté d'appréciation des magistrats et à l'impartialité des juridictions

et le tribunal d'instance et comporterait plusieurs sites, sous forme de chambres détachées, en dehors de son siège. Nous sommes opposés à la création de ces tribunaux, pour plusieurs raisons. sur un plan pratique, si l'objet de cet article est de favoriser l'égalité d'accès au service public de la justice, il nous semble que le cadre départemental n'est pas le plus approprié.

qui impose une affectation des dossiers selon des critères objectifs, des règles claires, précises, préétablies et stables, afin que le juge ne puisse être influencé par des éléments extérieurs.

Les chambres détachées seraient compétentes pour un certain nombre de contentieux de proximité, déterminés par décret en Conseil d'État, mais des compétences supplémentaires pourraient leur être attribuées sur décision des chefs de cour et sur proposition des chefs de juridiction., les chefs de juridiction décideront de la gestion des effectifs. Vous vous réjouissez, monsieur Bas, de la souplesse qui en résulterait dans l'affectation des magistrats et des fonctionnaires. Nous ne pouvons vous suivre dans cette appréciation, car ce mode de gestion mettrait à mal le principe d'inamovibilité du juge pour satisfaire l'objectif caché de pallier la pénurie des effectifs. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 10. La parole

présenter l'amendement n° 29 rectifié. Cet amendement vise à revenir sur la création de tribunaux de première instance uniques par département, en remplacement des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance. Il s'agit là d'un de nos principaux sujets de désaccord. Certes, des exceptions ont été prévues pour porter le nombre de tribunaux de première instance à deux dans certains départements, et l'on nous assure que les sites actuels permettront d'accueillir des chambres détachées. Cependant, nous ne sommes pas convaincus par l'argument

Les retours du terrain semblent montrer que les répartitions de compétences entre les tribunaux d'instance et les tribunaux de grande instance ne donnent pas lieu à de grandes difficultés. Certains professionnels ont également émis des doutes sur l'opportunité de créer des juridictions de très grande taille, plus difficilement pilotables. Il serait préférable de privilégier les structures moyennes. En outre, articulée avec la simplification de l'adaptation de la carte des implantations judiciaires prévue à l'article 17, cette réforme pourrait à terme aggraver l'enclavement des territoires les plus isolés de la République et réduire l'accès de certains justiciables au juge. Ce n'est pas acceptable pour nous ! Selon le rapport de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, déjà cité, la France figure parmi les onze pays européens étudiés où l'on trouve le moins de tribunaux par nombre d'habitants, alors que son territoire est le plus vaste de l'Union européenne. C'est bien la preuve que notre maillage juridictionnel territorial, déjà très distendu, ne doit pas être réformé dans le sens proposé.

Gouvernement ? Dans le cadre des chantiers de la justice, j'ai souhaité mettre en place un chantier spécifique dédié à l'adaptation de notre réseau des juridictions.

On ne peut nier que certaines matières juridiques sont devenues extrêmement complexes et ne peuvent plus être traitées occasionnellement par un juge moins spécialisé qu'un autre. C'est sans doute aussi

développé notre réflexion après une très large concertation et de nombreuses auditions. Il nous a semblé que la notion de tribunal de première instance présentait de très nombreux avantages, à commencer par celui de la proximité

reposant soit sur l'importance du litige en termes monétaires, soit sur les matières.

Nous affirmons de la manière la plus nette, nous écrivons dans notre texte qu'il ne s'agit pas de remettre en cause une seule implantation de tribunal.

La proximité, la lisibilité, la facilité d'accès, la qualité de gestion : tout commande de mettre en place le tribunal de première instance ! Les textes dont

Cet amendement de repli vise à supprimer le principe d'un tribunal de première instance par département et à compléter les critères d'implantation à prendre en compte. En plus de l'importance démographique et de la configuration géographique, critères déjà mentionnés à l'alinéa 13

par mes collègues. Quel est l'avis de la commission ?

L'expérimentation est d'ailleurs une démarche que le monde judiciaire connaît très bien, puisqu'il la pratique régulièrement et avec succès. On peut citer l'exemple récent du service d'accueil unique du justiciable, expérimenté entre 2014 et 2016. Cette expérimentation réussie permet aujourd'hui une entrée en vigueur progressive du dispositif dans les meilleures conditions.,

Madame la sénatrice, je tiens à vous redire que le Gouvernement est très attaché à ce que la question foncière en Polynésie puisse être réglée

Le scrutin est ouvert.

de la compétence du juge chargé des contentieux de proximité ». À ce titre, il est prévu que, en cas d'échec de la conciliation, le conciliateur pourra transmettre au juge le bulletin de non-conciliation, accompagné de sa proposition de règlement du litige, dans le respect du secret des échanges qui ont eu lieu au cours de la conciliation. Le juge statuerait alors sans entendre les parties, sauf s'il l'estime nécessaire ou si les parties le lui demandent. Bien sûr, nous considérons que les modes alternatifs de règlement des litiges permettent, le plus souvent, l'exercice d'une justice de qualité et l'apaisement des conflits. Toutefois, comme nous l'avons rappelé à plusieurs reprises au cours de ce débat, ces modes alternatifs ne doivent pas être pensés comme une solution à l'engorgement des tribunaux. Surtout, la proposition qui nous est faite ici, et qui montre une profonde méconnaissance à la fois du rôle du conciliateur et de celui du juge, heurte de plein fouet l'un des piliers de notre droit, à savoir le principe du contradictoire. Cela revient, en cas d'échec de la conciliation, à ériger le conciliateur en juge du fond, qui se déterminerait sur la base d'échanges confidentiels et dont les conclusions pourraient être homologuées sans aucun débat par le juge.

L'avis de la commission est défavorable. Je crois qu'il y a une incompréhension de ce qui est proposé. Je rappelle que la rédaction initiale prévoyait la possibilité en toute circonstance, pour les conciliateurs, de faire une proposition de règlement au juge.

et, le cas échéant, de lui fournir des informations utiles à la résolution du litige, voire de faire une proposition de règlement de celui-ci. Dans ce cas-là, aux fins d'accélérer le cours de la justice, le juge pourrait prononcer sa décision au vu de ce que propose le conciliateur,

Désormais, il s'agit de permettre aux conciliateurs de justice ayant tenté de concilier des justiciables après avoir été désignés par un juge de lui adresser une proposition de règlement du litige sur laquelle celui-ci pourrait statuer sans avoir systématiquement entendu les parties. Il faut bien entendu être extrêmement prudent avec les entorses au contradictoire et voir si elles sont véritablement justifiées, puisque les parties qui n'ont pas trouvé un accord devant le conciliateur voudront vraisemblablement s'en expliquer devant le juge. Cependant, la proposition qui est ici faite me semble extrêmement intéressante.

: La parole est à Mme Maryse Carrère. Cet amendement vise à supprimer la possibilité, pour les juges, de déléguer leur mission de conciliation à des assistants de justice. Il faut rappeler que, contrairement aux règles prévues pour les conciliateurs, qui doivent avoir exercé pendant trois ans dans le domaine juridique, aucune expérience n'est requise pour exercer la mission d'assistant de justice, qui reste par ailleurs assez vague- nous y reviendrons. Nous considérons que cette disposition nuit donc à l'esprit du recrutement d'assistants de justice, qui s'oriente vers des étudiants très qualifiés, désireux de se placer dans une situation d'apprentissage, dans la perspective de la préparation des concours du ministère de la justice. La faible rémunération de leur mission constitue en fait souvent un complément au financement de leurs études. C'est pourquoi il est important de maintenir cette relation d'apprentissage entre les magistrats et les assistants, plutôt que de placer ceux-ci dans une situation de délégation, pour des missions qui, par ailleurs, ne constituent pas le coeur de l'office du juge. Quel est l'avis de la commission ?

En cohérence avec l'amendement précédent, il est proposé d'étoffer le statut des assistants de justice. Pour le moment, il s'agit essentiellement de décrire les missions susceptibles de leur être confiées, toujours dans une perspective d'apprentissage. En effet, nous considérons qu'il est nécessaire de fixer certaines règles pour maintenir la qualité de leur accueil au sein des juridictions et s'assurer qu'ils ne soient pas simplement recrutés pour pallier le manque de magistrats et de greffiers. À plus long terme, nous pourrions réfléchir à l'établissement d'une passerelle vers l'École nationale de la magistrature pour les assistants de justice donnant satisfaction, en s'inspirant de celles déjà ouvertes au profit des juristes assistants et des professionnels du droit. Quel est l'avis de la commission ?

devenir itinérants pour pallier le défaut d'attractivité des professions judiciaires. Le tribunal de première instance, transformé en chambre détachée, ne peut quant à lui être déplacé au gré des politiques. C'est pourquoi nous sommes opposés à cette idée d'une révision périodique de la carte judiciaire.

Enfin, une refonte du réseau judiciaire, me semble-t-il, ne peut être envisagée qu'au regard d'un certain nombre de critères très objectifs liés à des évolutions procédurales et à des évolutions numériques ne présentant aucun caractère quinquennal.

Mme Josiane Costes. L'article 17 prévoit une procédure simplifiée pour réviser la carte judiciaire, reposant sur les observations des premiers présidents des cours d'appel et des procureurs généraux des ressorts. Les rapporteurs y ont ajouté la consultation des conseils départementaux. Afin que ces observations puissent être comparées d'un ressort à un autre, nous avions jugé utile de préciser dans la loi qu'elles reposent sur des données statistiques collectées selon des critères harmonisés. Il existe en effet différentes façons de comptabiliser les dossiers suivis par juridiction, ce qui pourrait biaiser les décisions d'implantation judiciaire. Quel est l'avis de la commission ?

l'exception des situations de surendettement, de la saisine du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants, par exemple. Je rappelle que cette contribution, ce droit d'ester avait été créé pour assurer le financement de la réforme de la garde à vue à laquelle avait été contraint le gouvernement de M. François Fillon. Fillon. Elle a été supprimée par la loi de finances pour 2014 sur proposition de Mme Taubira, alors garde des sceaux, au motif qu'elle constituait un véritable frein à l'accès au droit. Pour compenser la perte de recettes, une dotation budgétaire avait été créée. La présente

L'article 18 de la proposition de loi vise à rétablir la contribution pour l'aide juridique supprimée par la loi de finances du 29 décembre 2013. Elle serait désormais modulée, de 20 à 50 euros, en fonction du type d'instance engagée. Malgré les exemptions prévues pour les litiges prud'homaux et pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, cette mesure nous paraît, encore une fois, participer d'une vision comptable de la justice, dont les « usagers » devraient participer à la couverture du coût de fonctionnement. L'accès au droit, au juge, cela n'est plus à démontrer, est un problème majeur dans notre pays. Cette taxe constituerait un obstacle supplémentaire pour les plus fragiles de nos concitoyens. La justice de notre pays est exsangue, le manque de moyens humains et matériels est criant, et ce à tous les niveaux. Mais que nous est-il proposé ici ? De faire porter l'effort sur les plus précaires. Nous demandons la suppression de cette disposition, comme nous demanderons celle de l'article 19, qui rend obligatoire la consultation d'un avocat avant toute demande d'aide juridictionnelle. Investir dans la justice de notre pays ne doit pas se réduire à construire des prisons. Il est urgent de donner aux juges, aux greffiers et à tous les acteurs judiciaires les moyens de mener convenablement leurs missions.

Nous considérons que la réintroduction d'une contribution constituerait une régression, à rebours du principe de gratuité de la justice érigé dès la loi des 16 et 24 août 1790. En outre, cette contribution, dont le produit est affecté au Conseil national des barreaux, instaure un régime de financement des frais de justice excessivement complexe et difficilement compréhensible pour les justiciables.

D'une part, elle permet d'assurer un financement plus pérenne de l'aide juridictionnelle. D'autre part, cette contribution constitue, d'une certaine manière, manière, un instrument de régulation contre les recours abusifs. Enfin, elle connaît un certain nombre de dérogations qui viennent en atténuer la portée. Toutefois, nous considérons qu'une telle contribution

En revanche, une mission de deux mois va être confiée à l'Inspection générale des finances et à l'Inspection générale de la justice,

exemptées les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Nous considérons en effet qu'il n'est pas sain de créer un système à deux vitesses, où les uns auraient l'impression de contribuer deux fois au financement de la justice, en tant que contribuables puis en tant que justiciables que justiciables le droit de timbre, et les autres bénéficieraient de la solidarité nationale l'aide juridictionnelle et seraient exemptés de la contribution. Dans l'hypothèse malheureuse d'un rétablissement de la contribution, il nous paraîtrait plus juste que chacun paie à hauteur de ses moyens. par mes collègues. Quel est l'avis de la commission ?

Cette mesure nous semble porter atteinte au principe d'accessibilité de la justice que vise précisément à défendre cette proposition de loi, en introduisant un obstacle supplémentaire dans le parcours du justiciable qui souhaite saisir la justice mais n'en a pas les moyens.

relative à l'aide juridique, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé : « -Toute demande d'aide juridictionnelle est précédée de la consultation d'un avocat. Celui-ci vérifie que l'action envisagée n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. Cette consultation n'est pas exigée du défendeur à l'action, de la personne civilement responsable, du témoin assisté, de la personne mise en examen, du prévenu, de l'accusé, du condamné et de la personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. « La rétribution due à l'avocat pour préalable de culpabilité. « La rétribution due à l'avocat pour cette consultation est prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle si le demandeur remplit les conditions pour en bénéficier, à l'exception de celles fixées à l'article 7. « Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application

L'utilisation de la visioconférence est possible dans de nombreux cas, mais, pour certains d'entre eux, il convient d'obtenir l'accord de l'ensemble des parties ou du détenu. Un détenu peut donc aujourd'hui s'opposer à l'utilisation de cette modalité technique, par exemple pour sa comparution devant le tribunal correctionnel ou pour une audience au cours de laquelle il doit être statué sur son placement en détention provisoire ou la prolongation de sa détention provisoire. Sans remettre en cause le droit d'accès au juge, il est proposé de pouvoir recourir à la visioconférence dans l'ensemble des cas prévus aujourd'hui par la loi sans qu'un détenu puisse s'y opposer. Je tiens à rassurer la commission des lois : je ne propose aucune modification des cas prévus par la loi, notamment en matière pénale. Cette simplification permettrait de répondre en partie aux nombreux dysfonctionnements constatés en matière d'extractions judiciaires depuis l'extension de leur prise en charge par l'administration pénitentiaire. La correction de la réforme des extractions judiciaires figure en annexe à la proposition de loi. Il s'agit là, madame la garde des sceaux, d'un véritable fiasco. Dans certaines juridictions, plus de 50 % des extractions judiciaires ne sont pas exécutées, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner pour la suite de la procédure.

En matière pénale, de surcroît en matière de comparution personnelle devant le tribunal correctionnel, ne pas comparaître ou le faire par voie de visioconférence nécessite impérativement l'accord de la personne concernée. Si cet amendement était adopté, son accord ne serait plus nécessaire, ce qui constituerait, en matière pénale, une atteinte réelle à un droit

dénonce la lourdeur de la charge de travail, notamment de celle des missions non assumées. En effet, on ne trouve aujourd'hui aucun domaine touchant de près ou de loin la justice dans lequel un rôle ne soit réservé au ministère public. Pour certaines attributions, c'est un simple avis qui est demandé au parquet, mais, parfois, c'est également l'instruction complète du dossier et son suivi, alors qu'à l'évidence une autre autorité serait mieux placée pour y procéder. Le « livre noir » dresse ainsi une liste des attributions pour lesquelles l'intervention du parquet est dépourvue de sens réel et qu'il conviendrait donc d'assouplir. Si un grand nombre d'allégements nécessitent des modifications réglementaires,

question des moyens financiers et humains nécessaires au redressement de la justice, il convient également de s'attaquer à l'allégement des charges inutiles. À mon sens, le Gouvernement ne peut qu'accepter cet amendement de bon sens ! Quel est l'avis

L'instauration de la fonction de procureur général de la Nation permettrait de garantir une véritable indépendance de la justice en régulant les liens entre le pouvoir politique et le parquet.

que vous appelez de vos voeux. Je dois cependant rappeler que nous nous inscrivons pleinement, bien qu'un dialogue doive encore être noué avec l'ensemble des personnes intéressées à cette révision constitutionnelle, dans le cadre de l'article 20 de la Constitution, selon lequel « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation

pour présenter l'amendement n° 9. Dans l'état actuel du droit, les condamnations à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans, ou à un an si le condamné est en récidive légale, ne peuvent être exécutées sans le préalable obligatoire d'un examen de la situation du prévenu par le juge de l'application des peines, chargé de définir les modalités d'exécution de la peine. Considérant que ce dispositif a « « dénaturé le sens de la peine d'emprisonnement », les auteurs de la proposition de loi en demandent, au travers de l'article 27, la suppression.

Ces différents acteurs ont évoqué la nécessité d'établir un véritable bilan de l'application de la loi de 2009, qui est à l'origine de ce dispositif. Tous ont dit l'urgence de renforcer les moyens des juges de l'application des peines, certains ont regretté ce qu'ils considèrent comme une régression dans l'évolution du droit de la peine. Nous partageons leurs préoccupations, leurs revendications et demandons, en conséquence, la suppression de ces dispositions. Contrairement à vous, monsieur le président Bas, nous ne considérons pas que la seule peine qui vaille soit l'incarcération effective. Bien au contraire, l'emprisonnement, la désinsertion, la surpopulation carcérale sont autant de facteurs de récidive. Or la peine doit permettre au condamné de reprendre, à l'issue de celle-ci, toute sa place dans notre société. C'est pour cela qu'elle doit être le plus individualisée possible et qu'il faut donner aux juges les moyens pour ce faire. Par ailleurs, permettez-moi de vous rappeler que, notre pays étant loin de garantir la dignité de ses détenus, adopter des mesures qui auront pour conséquence une aggravation

Cet article va même plus loin : il abaisse le seuil de la peine pouvant être aménagée de deux ans à un an, et d'un an à six mois pour les condamnations en récidive.

faisant en sorte que le droit puisse être appliqué dans de bonnes conditions. En l'absence d'aménagement par la juridiction, la peine de prison sera mise à exécution sans que la situation personnelle du condamné soit examinée de manière approfondie.

Enfin, comme les rapporteurs- sur ce point, j'approuve leurs conclusions -, je regrette que les juridictions de jugement ne s'intéressent qu'insuffisamment à l'exécution effective des peines qu'elles prononcent, alors même que leur rôle ne se limite pas à la déclaration de culpabilité : il doit inclure

Je suis, au contraire, partisan de la diversification des peines et de leur adaptation, à la fois à la gravité des délits et des crimes commis et à la personnalité

Il faudra s'interroger sur les raisons de cette situation. En ce qui me concerne, madame Benbassa, je ne suis pas partisan de la peine de prison systématique. J'ai conscience, comme vous et comme toutes les personnes de bonne foi, que la prison n'est pas forcément la meilleure solution pour protéger

condamnées à des peines de prison ferme seraient en attente d'une décision du juge de l'application des peines. Ce n'est pas normal ! Le Président de la République lui-même, dans son projet présidentiel, a fait de cette

ou le sursis avec mise à l'épreuve, ou la contrainte pénale, si elle peut être mise en oeuvre, ou l'un des autres dispositifs en vigueur. Nous avons donc encore du chemin à parcourir.

a été instauré pour prévenir la récidive et pour seconder les efforts de réinsertion sociale par des injonctions de soins ou des mesures d'assistance. C'est une peine complémentaire

la proposition de loi vise à faire du suivi socio-judiciaire une peine complémentaire de portée générale susceptible d'être prononcée pour tous les délits et les crimes, afin de soumettre tous les condamnés, une fois leur peine d'emprisonnement purgée, à des obligations particulières pendant une certaine durée. Cette disposition nous paraît inutile, dans la mesure où un accompagnement est toujours possible

a maintenu l'interdiction des droits civiques résultant d'une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant le 1 mars 1994. Il en découle que les effets des incapacités de plein droit antérieures au 1 mars 1994 peuvent se poursuivre encore aujourd'hui. Permettez-moi, mes chers collègues, de prendre un exemple concret pour illustrer mon propos. Quelque temps avant l'élection présidentielle de 2012, M. Delvigne sollicite son inscription sur les listes électorales de sa commune.

les faits, alors qu'il a purgé sa peine et retrouvé une vie paisible, M. Delvigne est toujours privé de ses droits civiques.

Au-delà de ce cas particulier, ce sont des milliers de nos concitoyens qui sont aujourd'hui soumis à une déchéance civique à vie. La Cour de à vie. La Cour de cassation préconisait dès 2008 l'abrogation de l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992. à voter cet amendement et, ainsi, à mettre fin à une inégalité de traitement entre personnes condamnées, fondée uniquement sur la date de leur condamnation. Quel

Cette possibilité est toujours ouverte pour les personnes ayant été condamnées définitivement par un tribunal avant 1994. La difficulté tient au fait que, depuis 2010, le Conseil constitutionnel a une position constante en la matière

du Gouvernement ? Madame Benbassa, il est vrai qu'il existe une différence de traitement, donc une inégalité, entre les personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la réforme du code pénal, intervenue le 1 mars 1994, et celles qui ont été condamnées après celle-ci. Les premières ont été automatiquement privées de leurs droits civiques lorsqu'elles étaient condamnées pour des crimes ou, pour les délits, à des peines d'un certain montant les secondes n'ont pu l'être que si la juridiction l'a expressément décidé. Le nouveau code pénal était, sur cette question comme sur un certain nombre d'autres, moins sévère que l'ancien et plus respectueux du principe d'individualisation des peines ; c'était sa caractéristique principale. Pour autant, il n'existait aucune autre solution que de prévoir que les interdictions des droits civiques résultant de plein droit des condamnations prononcées avant 1994 demeuraient applicables, comme l'a prévu l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal. Si cela n'avait pas été le cas, en effet, toutes ces personnes auraient immédiatement, en 1994, retrouvé tous leurs droits, avaient été condamnées pour les faits les plus graves, à l'encontre desquelles, sous l'empire du nouveau code, les juges auraient certainement prononcé la peine complémentaire d'interdiction de droits civiques. Il y aurait également eu une inégalité de traitement au bénéfice des personnes déjà condamnées, puisque celles-ci ne pouvaient évidemment pas être jugées une nouvelle fois, afin que soit ou non décidé de compléter leur peine par une interdiction expresse de leurs droits civiques. La question se pose toujours aujourd'hui. Si vous supprimez l'article 370, tous ces individus retrouvent immédiatement leurs droits civiques. condamnée, par exemple, pour viol et assassinat à la réclusion criminelle à perpétuité en 1993 et qui, bénéficiant d'une libération conditionnelle, serait élargie demain, pourrait donc être inscrite sur les listes électorales, voter et se présenter à une élection. une autre, qui aurait été condamnée à la même peine pour des faits exactement similaires à la fin de l'année 1994, donc sous l'empire du nouveau code, avec, comme c'est vraisemblable, une condamnation de la cour d'assises à la peine complémentaire de privation de ses droits civiques, ne bénéficierait pas d'une telle clémence. Bien évidemment, comme le précise l'article 370 et comme vient de le dire à l'instant M. le rapporteur, le maintien de ces interdictions n'est prévu que sous réserve de la possibilité, pour le condamné, de demander leur relèvement, en application de l'article 702-1 du code de procédure pénale, devant le tribunal correctionnel, ou la cour d'appel, qui a prononcé la condamnation initiale, ou bien devant la chambre de l'instruction si la condamnation émane de la cour d'assises. Si les faits sont anciens

prononcé une peine d'interdiction des droits. S'il estime que tel n'aurait pas été le cas, il accordera évidemment le relèvement. Il me semble donc que l'article 370 ne porte en rien atteinte aux exigences d'équité que doit respecter notre droit pénal

monsieur le président de la commission des lois, messieurs les corapporteurs, mes chers collègues, La justice va mal. La réforme de l'institution judiciaire et la mise à niveau de ses moyens sont une urgence pour notre État de droit. » Ces mots ouvraient l'exposé des motifs de la proposition de loi qui nous a réunis aujourd'hui. Je les partage tous. Je suis en revanche convaincue, comme l'ensemble des membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, que certaines des dispositions de ce texte, loin de participer au redressement de la justice, constituent une sérieuse remise en cause du fonctionnement de l'institution judiciaire et des principes fondateurs de notre droit. Nous considérons la question des moyens alloués à la justice comme un indispensable corollaire à son indépendance. Ceux-ci doivent être renforcés, mais certainement pas, comme vous nous le proposez, par une approche managériale et comptable de la justice. Consolider l'état de droit est, pour nous aussi, une priorité-nous avons d'ailleurs été bien seuls à le défendre lorsqu'il s'est agi de faire entrer les mesures de l'état d'urgence dans notre droit commun -, mais la réponse ne peut être uniquement répressive. Monsieur le président de la commission des lois, elle doit être pensée en termes de réhabilitation et de réinsertion. C'est bien l'humain qui doit être au coeur de notre politique pénale. cela non pas par angélisme, mais par pragmatisme. Nous le savons, le tout-carcéral, le tout-répressif, cela ne marche pas ! Cela ne fait pas diminuer le taux de récidive, cela ne porte pas ses fruits en matière de réinsertion De surcroît, nous ne cesserons de le rappeler, l'exigence de respect de la dignité doit être aussi considérée derrière les barreaux des prisons. L'incarcération ne doit pas valoir exclusion ; le détenu reste membre de la cité et doit donc conserver ses droits fondamentaux. Parce que ce sont ces valeurs et ces principes qui guident notre action politique, nous voterons contre ces propositions de loi. Personne ne

à juste titre, de mettre fin à la procédure de gel budgétaire pour les programmes des juridictions judiciaires et du Conseil supérieur de la magistrature, afin de sanctuariser les crédits consacrés au fonctionnement de l'autorité judiciaire. Nous souhaiterions aller plus loin, en ouvrant le débat sur l'opportunité de créer une nouvelle mission budgétaire, à côté de la mission « Justice », rassemblant les crédits consacrés à l'administration pénitentiaire.

qu'ils ont des ramifications communes. Cependant, il nous semble important de nous assurer que l'ambition de régulation de la population carcérale n'influence pas la décision des juges chargés de prononcer ou de faire appliquer des sanctions. De ce point de vue, une plus stricte séparation budgétaire nous semblerait salutaire. Cette séparation pourrait ainsi distinguer les deux fonctions qui cohabitent actuellement au sein de la mission « Justice » : juger et punir. Enfin, nous souhaiterions insister sur le fait que des marges de manoeuvre existent. Certains observateurs avisés ont fait remarquer que, dans la période courant de 2002 à 2016, les crédits accordés aux juridictions judiciaires ont augmenté de 60 %, contre 109 % pour les juridictions administratives. Il est grand temps de traduire ces constats en engagements réels et de prendre des mesures budgétaires à la hauteur des difficultés de fonctionnement que rencontre l'autorité judiciaire. Quel est l'avis de la commission ?

Comme le relèvent l'ensemble des magistrats, il ne convient pas d'inscrire ce principe dans la loi, car cela interdirait toute exception due à des circonstances particulières, comme une maladie, par exemple. En outre, cette solution autoritaire aurait pour effet, ainsi que le soulignent les magistrats, de renforcer encore la désaffection pour les juridictions dites « fragiles » et peu attractives, les magistrats craignant de devoir y rester trois ou quatre ans. La conséquence serait la multiplication des demandes de disponibilité, lesquelles apparaissent bien souvent comme la seule solution pour quitter une affectation devenue insupportable. S'il est vrai que certaines fonctions ou juridictions sont en difficulté, car elles sont délaissées, le problème ne sera résolu que par une gestion plus adaptée des ressources humaines par le ministère de la justice. C'est ainsi qu'une plus grande stabilité des magistrats dans leur poste sera possible. Quel

S'agissant de la difficulté, pour certaines juridictions, d'accueillir du monde, il est vrai que, aujourd'hui, la vacance des postes est telle que des magistrats sont tentés de partir très vite vers des emplois qui leur conviennent mieux que ce qu'ils acceptent en première affectation.

Ce délai est porté à trois ans pour les emplois de chefs de juridiction et de cour. Il nous semble donc que la fixation, dans l'ordonnance statutaire, d'une durée minimale d'exercice des fonctions n'est pas nécessaire et pourrait, au contraire, emporter des conséquences néfastes pour le corps des magistrats sur l'ensemble du territoire. En effet, le défaut d'attractivité de certaines juridictions et de certaines fonctions risquerait d'être accru si les magistrats y sont nommés pour une durée incompressible de trois ou quatre ans. Nous ne le souhaitons pas, parce que cela aboutirait à la suppression d'une indispensable souplesse dans la gestion des ressources humaines,

pour les conseillers ou avocats généraux référendaires à la Cour de cassation, et de sept ans pour les chefs de cour et de juridiction. Ce dispositif apparaît suffisant et adapté pour assurer la mobilité des magistrats et amoindrir les effets négatifs d'un exercice professionnel trop long dans une même juridiction. Cette mesure risque de créer des difficultés de gestion en cas d'élargissement à toutes les fonctions de magistrats. C'est la raison pour laquelle je suis favorable à l'amendement proposé. Je mets

sauf exception prévue par ailleurs. Dans une perspective d'efficience, nous considérons que des gains de productivité pourraient être effectués en étendant cette obligation à la fonction, afin de permettre une plus grande spécialisation de nos magistrats. Il n'est pas rare, en effet, d'observer d'importantes rotations susceptibles de nuire à la continuité du service. Quel est l'avis de la commission ?

commission, modifié, l'ensemble de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Le scrutin est ouvert.

Merci